L'ordre du jour appelle le débat sur les initiatives européennes en matière de simplification et d'allègements de la charge administrative pesant sur les entreprises. Ce débat a lieu à la demande du groupe Les Républicains. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté, si le juge nécessaire. de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes, Madame la Ministre. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, et ce pour une minute. Madame la Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce départ, Monsieur Jean-François Rapin, pour le groupe Les Républicains, et ce pour huit minutes. À vous, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie le groupe Les Républicains qui a souhaité ce débat sur les initiatives européennes en matière de simplification et d'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises. Ce débat intéresse au-delà de nos murs. Une contribution m'a ainsi été adressée par le Conseil national des barreaux qui souligne les enjeux de sécurité juridique et de cohérence du marché unique liés aux initiatives actuellement prises par la Commission européenne. Il y a quelques semaines, conjointement avec la délégation aux entreprises, la Commission des affaires européennes a organisé une table ronde sur la simplification. Elle a également adopté une proposition de résolution européenne que j'ai présentée avec le président Ritman pour défendre la reconnaissance par l'Union européenne des entreprises de taille intermédiaire. Lors de notre réunion conjointe, les représentants des entreprises nous ont fait part de leur vive préoccupation quant à la mise en œuvre de plusieurs réglementations européennes, mais ils ont aussi souligné un changement d'approche de la nouvelle Commission européenne. Soyons clairs, cette nouvelle approche, dont la restauration de la compétitivité européenne est l'un des maîtres mots, répare certaines erreurs commises sous la précédente mandature. La période 2019-2024 a en effet été marquée par des mesures fortes et parfois très symboliques de régulation de certains pans de notre économie. Je pense évidemment aux règles adoptées en matière de durabilité de devoirs de vigilance, les fameuses CSRD, CS3D que la Commission européenne propose désormais de réviser. Je pense aussi aux paquets ajustements à l'objectif 55 qui a posé des règles à certains égards trop contraignantes, et nous l'avons souvent dit ici pour notre industrie, comme l'avait souligné le Sénat, dont la fin des véhicules thermiques neufs en 2035, jusqu'aux modalités de la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que la Commission européenne envisage désormais de reprofiler, et je m'en félicite. La Commission européenne semble ainsi s'engager dans une nouvelle voie, plus réaliste et plus en phase avec les contraintes des entreprises. Plus consciente aussi, me semble-t-il, du basculement auquel nous faisons face au niveau mondial. L'Union européenne fait face à des stratégies économiques très agressives de la part de nombreux concurrents, en particulier bien sûr la Chine et les États-Unis. L'administration Trump se montre aujourd'hui particulièrement véhémente, mais nous ne devons nous ne devons pas oublier que c'est l'administration Biden qui a fait adopter l'Inflation Reduction Act. Confrontée à cette situation, l'Union n'a pas d'autre choix que de devenir plus productive, de libérer son potentiel d'innovation, de simplifier et de redonner de la cohérence à sa réglementation. Mario Draghi souligne avec force que sans un effort de productivité, l'Europe ne pourra pas, ne pourra pas, et je le cite, être à la fois un leader des nouvelles technologies, un phare de la responsabilité climatique, et un acteur indépendant sur la scène mondiale. Elle ne pourra pas non plus financer son modèle social et elle devra revoir à la baisse certaines de ses ambitions, si ce n'est pas toutes. La Commission européenne a ainsi présenté fin janvier une ambitieuse boussole pour la compétitivité qui passe en particulier par un choc de simplification pour les entreprises, c'est-à-dire un allègement des contraintes administratives qui pèsent sur elles. Selon la Commission européenne, cette fois-ci, nous sommes sérieux. L'ambition est forte, je m'en fie ici, puisqu'elle vise à réduire d'au moins 25% la charge administrative qui pèse sur les entreprises et d'au moins 35% celle qui pèse sur les PME. Mais à quoi nos entreprises peuvent-elles s'attendre en pratique après plusieurs années pendant lesquelles elles se sont vues imposer des contraintes nouvelles ? Que les choses soient claires, loin de moi l'idée qu'il faille rejeter en bloc la réglementation fixant les obligations aux entreprises en matière de durabilité ou de responsabilité sociale et environnementale, rappelons qu'avant la CSRD, en 2014, la directive NFRD avait déjà imposé à plus de 11 000 entreprises de réaliser leur reporting extra financier. La Commission européenne ne propose pas de déréguler, c'est un autre débat, mais de simplifier et il y avait urgence tant s'agissant du périmètre des entreprises couvertes que du nombre des indicateurs que les entreprises devront fournir. On avait mis en place une véritable usine à gaz. Je ne perds pas non plus de vue l'enjeu de la transition écologique, mais nous devons être lucides et responsables. Les entreprises européennes sont de très loin parmi les plus vertueuses du monde sur le plan écologique et social. dans un contexte de concurrence exacerbée, ne leur imposant pas de contraintes excessives qui vont les conduire à s'implanter en dehors de l'Union ou qui vont favoriser leurs concurrents bien moins vertueux. Je me réjouis donc de l'adoption rapide de la directive dite Stop the Clock, qui a retardé de deux ans la mise en œuvre de la directive sur la durabilité et d'un an celle de la directive sur le devoir de vigilance. Il faut maintenant réviser le fond de ces dispositifs et veiller à une réelle cohérence de l'ensemble des normes au niveau européen. Je pense notamment à la taxonomie, mais aussi à une bonne articulation entre le droit national et le droit européen. Je ne m'y connais pas non plus les craintes exprimées par le Conseil national des barreaux. En matière de durabilité, la France, en transposant la directive la première dès 2023, fait figure de bon élève. Arrêter la pendule permettra de donner aux entreprises concernées le temps de s'adapter. Mais qu'en sera-t-il de celles qui ont déjà scrupuleusement rempli leurs obligations ? Comment éviter une forme de prime aux mauvais élèves ? S'agissant du devoir de vigilance, nous avions déjà alerté sur le poids de la charge pesant sur les entreprises pour s'assurer du respect des normes en matière de droit de l'homme et de protection de l'environnement tout au long de la chaîne de valeurs. Là encore, nous ne pouvons que nous féliciter de l'allègement proposé, notamment en concentrant les mesures de vigilance aux seuls partenaires directs et en diminuant la fréquence de déclaration qui incombe aux entreprises. les entreprises ne seront-elles pas soumises à des obligations de reporting différentes, selon que leur chaîne de valeur est composée d'un grand nombre de petites entreprises ou, principalement, d'entreprises de plus grande taille. J'observe que le nouveau gouvernement allemand devrait proposer d'abroger la loi sur les obligations de devoir de vigilance dans les chaînes de valeur entrées en vigueur en janvier 2023 pour la remplacer par la loi sur la responsabilité internationale des entreprises qui mettra en œuvre la directive européenne au cours de la renégociation. En attendant, il n'y aura pas de sanction pour les entreprises qui ne respecteraient pas la loi actuellement en vigueur à l'exception des violations massives des droits de l'homme. Il est donc urgent d'adopter le premier train de simplification contenu dans le paquet Omnibus du 26 février pour éviter toute distorsion de concurrence au sein de l'Union. Je veux également souligner l'intérêt que pourrait présenter la proposition de création d'un 28e régime juridique. Il se veut le moyen pour les entreprises innovantes de bénéficier d'un ensemble de règles uniques lorsqu'elles investissent et exercent leurs activités, ou que ce soit au sein du marché unique. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner des précisions quant à la position du gouvernement sur ce dossier ? Au-delà de ces premières mesures, il est nécessaire que la démarche de simplification se poursuive dans la durée. D'autres paquets de simplification sont attendus en faveur des ETI, mais aussi pour redonner de l'air au secteur agricole qui a été si contraint ces dernières années. Nous avons besoin de redonner de la compétitivité aux entreprises dans l'ensemble des secteurs économiques, Nous avons besoin de mieux prendre en compte leur capacité à absorber les normes en traitant en particulier de manière adaptée les PME et les ETI, mais aussi de mieux prendre en compte leur capacité à faire face à la concurrence internationale. Pouvez-vous Madame la Ministre, affirmer devant nous la détermination du gouvernement à défendre cette démarche de restauration de la compétitivité ? Pouvez-vous également nous préciser les mesures que vous soutenez plus particulièrement ainsi que vos éventuelles lignes rouges ou mise en garde. Je vous remercie. Merci. Merci. Madame la Ministre, vous souhaitez intervenir maintenant. Madame la Ministre Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'Intelligence Artificielle et du Numérique. Allez-y, Madame la Ministre. Vous intervenez en début de débat, donc vous n'aurez pas besoin de conclure. Monsieur le Président, Monsieur le Président Rapin, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce débat sur les travaux européens en matière de simplification des obligations administratives de nos entreprises qui est une des priorités de l'action du gouvernement comme vous le savez

Par conséquent, en effet, monsieur le Président, permettez-moi de prendre le temps d'un petit propos liminaire qui sera gage de concision de la conclusion des débats. A la suite de la publication du rapport Draghi, Nous avons un constat unanime sur le déficit de compétitivité de l'Union européenne et la Commission, suite à ce rapport, a agi puisque dès fin février, elle a proposé un paquet omnibus de simplification de la réglementation en matière de durabilité pour commencer. Il ne s'agit en aucun cas, je tiens à être très claire au travers de cet omnibus, de remettre en question les objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne dans le cadre du Pacte vert, car ces objectifs sont eux-mêmes gages de compétitivité, ni sont leadership en la matière. Nous savons que l'inaction environnementale est un risque majeur. Selon le réseau des banques centrales sur le climat, la poursuite des trajectoires climatiques actuelles conduirait à une perte de 15 à 20 % du PIB mondial d'ici 2050. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Elle marque le premier dépassement du seuil des 1,5 degrés de réchauffement. Dans ce contexte, la mise en œuvre des objectifs du Pacte vert reste bien un apératif Pour autant, pour atteindre ces objectifs, les entreprises doivent pleinement intégrer leurs impacts et les risques environnementaux dans leur gestion stratégique sans perdre en compétitivité. En pratique, ces enjeux deviennent constitutifs de relations d'affaires tandis que les institutions financières les intègrent de plus en plus dans leurs décisions d'investissement. Il est décisif de s'appuyer sur l'expérience concrète de nos entreprises européennes dans un contexte où certaines grandes puissances se désengagent politiquement de cette lutte contre le changement climatique. Pour atteindre les objectifs du Pacte vert, cependant, l'appel suite au rapport Draghi a bel et bien été entendu et la France prend toute sa part pour faire en sorte que notre réglementation soit proportionnée, ne pas freiner notre compétitivité. En ce qui concerne le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont vous avez parlé, le paquet Omnibus prévoit de limiter le mécanisme aux importations de plus de 50 tonnes de marchandises contre le seuil initial de 150 euros. C'est important de le mentionner parce qu'il s'agit d'une simplification massive efficace. Elle sort du champ 92% des entreprises mais couvre toujours 98% des émissions. Un exemple à suivre. Le paquet Omnibus révise également la directive CSRD qui requiert la publication d'informations auditées et comparables en matière de durabilité. Nous le constatons actuellement. L'exercice demandé par le CSRD est excessivement lourd. Le paquet Omnibus prévoit ainsi de recentrer la directive sur les entreprises de plus de 1000 salariés, ce qui conduit à excepter 80% des entreprises. Un décalage de deux ans du calendrier est aussi prévu, en particulier pour les entreprises non cotées. Enfin, le volume des informations à publier va être réduit. Il s'agit d'une simplification très forte que nous soutenons vivement. Au niveau national, nous avons pris le plus tôt possible, dans la loi d'adult il y a quelques semaines, des dispositions de transposition. s'agissant de la directive CS3D sur le devoir de vigilance, l'enjeu de négociation européenne et de simplifier la directive actuelle qui va au-delà de la loi française et d'assurer des conditions de concurrence équitables. La proposition de la Commission apporte des modifications bienvenues qui renforcent la proportionnalité du cadre, comme la focalisation des localisation des mesures de vigilance sur les partenaires directs. Le gouvernement est favorable à des modifications supplémentaires comme le rehaussement de seuils à 5000 salariés en cohérence avec la loi française afin de limiter son application aux plus petites entreprises ayant les moyens humains et financiers suffisants ainsi qu'une influence véritable sur leur chaîne de valeur. Par ailleurs, la suppression d'un régime de responsabilité civile harmonisé se ferait au détriment des entreprises françaises. Constitue un point fort de la négociation actuellement menée. Comme vous le voyez, le travail de simplification ne recule pas devant l'obstacle. Le gouvernement agit avec détermination pour que cette simplification soit ambitieuse, adaptée aux réalités économiques, mais sans compromettre nos objectifs. Premier, j'insiste sur ce point. renforcer notre compétitivité en limitant la lourdeur administrative nous permettra d'atteindre de façon pragmatique les objectifs du pacte vert qui reste notre priorité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Là dans l'insuite du débat, la parole est à Monsieur Gérard Lailaig pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste Calaqui et ce pour cinq minutes à vos chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission européenne a donc présenté le 26 février dernier une proposition de directive dite Omnibus afin, je cite, de réduire les charges administratives et réglementaires pesant sur les entreprises et d'au moins 25 %. Sous prétexte de compétitivité, cette proposition fragilise plusieurs avancées récentes, la responsabilité sociale des entreprises, la finance durable et les exigences accrues de transparence. Or, nos entreprises sont dans une situation compliquée parce que l'économie contemporaine est régie par une forme de prime ovis. En gros, plus une entreprise a des pratiques délétères pour l'intérêt général, plus elle sera profitable. Si vous décidez de délocaliser pour produire dans des pays où les normes sociales et environnementales sont limitées, vous obtenez des coûts de production moins élevés et vous êtes donc plus compétitifs. Forcément, pour les entreprises qui veulent produire en France localement tout en respectant le droit applicable, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. La pratique du fast fashion dans le textile est l'incarnation de ces pratiques délétères. Ces entreprises vendent à bas prix des produits fabriqués dans des conditions déplorables et acheminés souvent par avion. En face, des PME françaises qui veulent produire en Europe du textile qualitatif sont étranglés par cette concurrence déloyale. Aujourd'hui, avec la guerre commerciale qui a été engagée par Donald Trump, le phénomène pourrait s'amplifier. L'afflux de produits chinois appricassés qui ne trouvent plus de débouchés aux États-Unis vont investir le champ européen et c'est déjà notamment le cas des voitures électriques. Les entreprises de plusieurs secteurs ont donc besoin de régulation pour être protégées de ce système pernicieux. Et je prends, par exemple, la loi anti-fast fashion qui avait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2024. Elle propose notamment d'augmenter les contributions financières payées par ces entreprises dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, prenant en considération l'impact environnemental des produits mis sur le marché. ce type de mesures participeraient à réduire la concurrence déloyale que subissent nos acteurs du Made in France ou du Made in Europe. Méfions-nous donc de certaines préconisations qui affirment que la régulation est un fardeau administratif, elle serve des intérêts prévus et ses lobbies profitent des inquiétudes sur le commerce international pour remettre en cause tout le cadre réglementaire. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents dans certains carrefours qu'il faut pour autant supprimer les feux rouges. C'est au contraire, en régulant la vitesse et le trafic, qu'on peut fluidifier la mobilité. Les entreprises ont besoin de régulations qui les protègent, du dumping social et environnemental. Sans régulation, c'est toujours la loi du plus fort et du moins scrupuleux qui s'applique. L'Europe fait face à une perte de souveraineté économique. Si l'on veut s'en sortir, on a tout intérêt à préserver la qualité de nos emplois, notre système de santé, nos sols, la qualité de l'air et de l'eau. Et pour ça, il faut des règles. L'Europe a la possibilité d'incarner une autre économie sociale et écologique. C'est aussi ce qui lui permettra de rester une puissance durable sur la scène mondiale. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie d'avoir porté notre attention sur un certain nombre de points. Avant de revenir sur les points sur la fast fashion et sur les produits chinois sur lesquels nous avons été particulièrement occupés avec les ministres de Bercy ce matin, peut-être vous rejoindre sur le fait que, oui, nous entendons beaucoup parler de cette Europe qui régule. Et je crois que c'est très juste, nous devons faire la différence entre l'objectif de la régulation, qui très souvent en Europe est un objectif de protéger nos valeurs et la manière dont nous voulons que notre union fonctionne, et l'application de cette régulation sur laquelle nous sommes bien sûr à la tâche d'avoir le plus de simplification possible pour ne pas ralentir nos entreprises qui elles-mêmes sont porteuses de ces valeurs. Donc il ne faut pas se laisser enfermer dans ce discours qui est parfois instrumentalisé, je vous rejoins là-dessus, sur le fait que la régulation est une fin en soi et ne serait que mauvaise. Sur la partie fast fashion et produits chinois, deux choses. La loi anti fast fashion que vous avez mentionnée arrive dans votre hémicycle très prochainement, je crois le 2 et 3 juin, et donc ça va étudier ici, c'est une bonne chose et nous serons très attentifs à l'évolution des débats parce que le risque que vous mentionnez. Je l'ai vu de mes propres yeux ce matin autour du ministre Éric Lombard. Nous étions réunis avec la ministre Amélie de Montchalin et la ministre Véronique Louvagie pour à Roissy voir cet afflux de petits colis, les colis en dessous de 150 euros, qu'achètent nos concitoyens par centaines de millions, 800 millions de colis chaque année et qui aujourd'hui présentent des risques avérés, on a beaucoup discuté avec les douanes et les différents services qui étaient présents, des risques d'abord pour les français parce que 94% de ces colis ne sont pas en conformité, des risques pour notre économie, contrefaçon, ce genre de choses, et des risques aussi bien sûr pour nos finances publiques puisqu'ils ne sont pas toujours bien déclarés. Et donc nous allons renforcer les contrôles et madame la ministre Amélie de Montchalin a parlé du fait d'instaurer des frais de gestion pour couvrir ces contrôles car nos concitoyens ne payeront pas le prix de ces contrôles. Merci. Vous voulez reprendre la parole, M. Lelec ? Non, c'est bon. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Fernic du groupe écologiste Solidarité et territoire. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le paquet Omnibus proposé par la Commission européenne entend, prétend alléger les charges administratives pesant sur les entreprises. Je crois que derrière ce vernis de simplification, c'est en réalité un très net coup de frein à la transition écologique européenne qui se concrétise. On veut nous faire croire que l'objectif réel serait de faciliter la vie de nos entrepreneurs écrasés par les formalités administratives. On veut nous faire croire que les obligations sociales et environnementales seraient des tracasseries qui, permettez-moi l'expression, pourriraient la vie des acteurs économiques sans rien faire avancer. Je crois que parler en l'occurrence, quand on regarde le contenu de ce paquet Omnibus, De simplification, ça relève de l'abus de langage. Ce qui se joue réellement, ce n'est pas la suppression de l'ordre administrative. En vérité, c'est un renoncement. une régression par rapport à des avancées qui ne sont pas faites à la légère, à des avancées qui ont été concertées, négociées, des négociations de trilogues difficiles, ça a été fait en connaissance de cause, c'est l'acquis de la précédente législature du pacte vert. Et donc avec ce paquet omnibus, on a une régression. Et si notre Sénat devait abonder dans ce sens, ça serait aussi une régression pour notre Sénat. Parce que je me rappelle, c'est pas si loin, c'était en 2022 de la résolution européenne, résolution du Sénat, que je co-rapportais avec Christine Lavarde et Didier Marie, de façon transpartisane, sur la directive de devoir de vigilance. Je me rappelle des recommandations, c'était l'an dernier de la commission d'enquête sur les obligations de total énergie. Tout cela était exigeant, ambitieux pour la directive de devoir de vigilance dont Ce paquet Omnibus prône l'affaiblissement aujourd'hui. Je crois que c'est un choix politique, délibéré, porté, il faut le dire, par la droite et l'extrême droite européenne. Au prétexte d'une simplification, tout ce qui relève du progrès environnemental ou des droits sociaux à l'échelle de la planète est pris pour cible. Les règles de RSE sont pointées du doigt comme bouc émissaire. des difficultés des entreprises. Avec ce paquet Omnibus, quelques principaux reculs qu'on peut citer, ce serait le report dans le temps contre-productif pour la mise en oeuvre CSRD et Vigilance. Pour la directive CSRD, le champ d'application proposé à présent épargnerait 80% des entreprises qui auraient dû être assujetties. Cela ne concernerait en définitive que 0,02% des entreprises européennes. L'obligation d'évaluation des impacts négatifs de l'activité de l'entreprise ne se ferait plus régulièrement tous les ans mais tous les cinq ans. On supprimerait l'obligation de rompre les relations commerciales dans le cas d'incidence négative avérée. Le devoir de vigilance surtout ne s'appliquerait plus à toute la chaîne d'activité. C'est là le principe même de cette directive qui serait liquidée. Enfin, il y aurait perte de la possibilité du recours juridique pour les victimes. Madame la Ministre, chers collègues, je crois que quand on affaiblit les obligations de reporting, quand on lâche sur la régulation, on ouvre les vannes. au dumping social et environnemental. Et ce dumping, c'est précisément ce qui malmène nos entreprises. C'est précisément ce qui entrave la réindustrialisation aujourd'hui. Vouloir affaiblir nos instruments extraterritoriaux, pousser à l'adoption de ce paquet omnibus, s'est allé, il faut le dire, à l'encontre de nos objectifs de souveraineté industrielle. Notre pays, la France, a été pionnière du devoir de vigilance suite à l'effondrement du Rana Plaza. Nous étions à l'avant-garde. En sapant de cette façon nos conquis sociaux et environnementaux, on va perdre un temps précieux alors qu'ailleurs la résilience des entreprises se prépare. La Chine, et oui la Chine, nous talonne en matière d'exigence dans les standards de durabilité. L'Australie, le Japon, le Canada sont en train d'adopter des législations allant allant dans le sens du devoir de vigilance. Voulons-nous vraiment perdre notre avance ? Cette dérégulation se ferait au détriment de la souveraineté européenne, de l'emploi des entreprises qui ont investi, puisque revenir sur les règles déjà votées encourage le vice et sanctionne la vertu.

vous rappelez d'abord que l'objectif du Pacte vert, 55% de réduction des émissions d'ici 2035, est bien un objectif que nous maintenons avec détermination au niveau européen. Et s'il ne fallait citer que des arguments économiques, mais je l'ai bien sûr cité tout à l'heure, il ne s'agit pas uniquement d'arguments économiques, je l'ai dit dans mon propos liminaire, La trajectoire climatique actuelle nous mènerait à 15 à 20% d'impact sur le PIB mondial. La question de la simplification qui est en cours, c'est celle de trouver la simplification la plus utile, la plus intelligente pour continuer à avancer vers cet objectif mais sans alourdir la charge pour nos entreprises. J'ai donné l'exemple le plus parlant mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières qui, en retirant 92% des entreprises du champ, couvre toujours 98% des émissions. Vous avez parlé du devoir de vigilance. Je veux vous rappeler que notre position, et c'est une négociation avec plusieurs pays européens, mais la position de la France, la position du gouvernement français qui a été, vous l'avez bien dit, précurseur sur le devoir de vigilance, c'est bien de continuer à avoir un certain nombre d'obligations et notamment nous avons fait savoir que la suppression d'un régime de responsabilité civile harmonisé se ferait au détriment de nos entreprises françaises et c'est un point très fort de négociation pour nous. Nous y sommes particulièrement attentifs. Je sais que dans le paquet Omnibus actuel, il s'agit de toutes les réglementations qui concernent les devoirs de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Pour autant, Vous rappelez que nous sommes aussi au travail pour simplifier tous les différentes directives européennes, y compris les directives en cours comme FIDA au risque sur le secteur financier, sur lequel nous sommes aussi au travail. Et on parlait tout à l'heure du secteur du numérique. Le secteur du numérique aura son propre omnibus en octobre de cette année et nous travaillons à réfléchir aussi à la simplification sur ces questions. Donc toutes les les directives sont bien concernées. Si, chers collègues, vous ne souhaitez pas réintervenir, j'ai bien compris. La parole est maintenant à monsieur... donnant à M. Michael Weber, notre collègue du groupe socialiste, écologiste et républicain. A vous, chers collègues. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, face à une mondialisation sans foi ni loi qui creuse les inégalités et nous pousse vers un modèle de consommation toujours plus destructeur pour la santé humaine et l'environnement, la norme peut être protectrice. La déréglementation et la dérégulation financière sont une réponse dangereuse au haro contre la charge administrative. Un espace existe entre bureaucratie et réglementation nécessaire pour en diminuer la complexité sans restreindre nos exigences. La frontière est cependant ténue. L'Europe doit fonder sa compétitivité sur les atouts de son modèle social qui est unique au monde et ne rien renoncer de son ambition. Seule l'Europe porte aujourd'hui un projet et une vision cohérentes pour une économie responsable et durable. En ce sens, l'Union européenne réglemente l'accès à son marché pour favoriser le développement d'entreprises européennes vertueuses, pour limiter nos émissions de carbone, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et la pollution de l'air et améliorer notre alimentation. L'Europe met enfin en œuvre des mesures concrètes pour garantir le respect des droits humains, pour que nos valeurs ne deviennent pas seulement des idéaux vénérables inscrits dans nos Constitutions et un alibi juridique absent de nos vies quotidiennes. L'argument est aussi d'ordre économique. L'Europe propose un modèle de vie attractif et innovant, fondé sur la durabilité. Le renforcement de la qualité de nos modes de production et de consommation est l'avantage compétitif du modèle économique européen. Les investissements verts, l'innovation durable, l'harmonisation d'un marché européen qui pèse autant que celui des États-Unis sont ainsi des piliers d'une compétitivité européenne qui n'oppose pas la stabilité financière à la transition écologique et au respect des droits humains. Or, c'est au nom de cette même compétitivité que l'on veut aujourd'hui saper les avancées majeures de l'UE en matière de droits humains, d'environnement et de climat. Dans cette course aveugle à la compétitivité, comparant un instant nos modèles sociaux, L'espérance de vie en Europe est la plus élevée du monde et les inégalités y sont les plus faibles. Les émissions carbone sont trois fois plus élevées aux États-Unis qu'en Europe. La production d'électricité en Europe est la moins carbonée et atteint 45% en renouvelables alors que les États-Unis plafonnent à 15%. La surface agricole en bio est proche de 10% en Europe lorsqu'elle est de moins de 1% aux États-Unis. Le continent américain a triplé sa consommation de pesticides quand l'Europe l'a réduite de 5%. Les politiques que nous menons collectivement ont bel et bien des résultats concrets, mais nos engagements pour une économie durable et responsable suscitent des oppositions fortes de nos partenaires et concurrents internationaux. L'administration américaine, comme à l'époque de Kissinger, n'hésite pas à s'immiscer dans nos politiques pour les contourner, pour torpiller le pacte vert européen et défaire les ambitions agro-écologiques de l'Europe. Aux États-Unis, les normes et les fonds ESG sont pris pour cible depuis 2022. Le mot d'ordre semble pourtant être toujours plus de profit pour les grands groupes, plus d'énergie fossile, plus de ségrégation sociale, plus d'inégalité, de fraude, d'intimidation, de précarité et moins de droits humains, moins d'environnement, de solidarité et de justice. Cette politique unique et absurde est aujourd'hui présentée comme une recette payante, pas certaine dans une course à la croissance ou où la norme est perçue comme un obstacle. Subissant cette pression politique, la Commission européenne ouvre aujourd'hui la boîte de Pandore en voulant revenir sur ses normes les plus ambitieuses, en les reportant sinédiers ou en restreignant leurs champs d'application au risque de les vider de leurs substances et de ne produire que des coquilles vides. Or, ces retours en arrière, sous la pression internationale, ces va-et-vient incessants nous affaiblissent collectivement, créer de l'incompréhension et de l'instabilité dont les entreprises européennes sont les premières à souffrir. Je vous remercie. apporter votre éclairage. Allez-y. l'objectif de simplification qu'est celui de l'Europe, c'est trouver le bon équilibre entre eux, trop de bureaucratie, mais sans réduire notre ambition. Je l'ai redit tout à l'heure. vous avez parlé de vider de sa substance et je pense important de rappeler que avec CSRD dans la version actuelle, l'Europe reste leader, reste très ambitieuse, reste plus ambitieuse que des standards internationaux comme l'ISSB que nous connaissons bien par l'implication de certaines personnes qui est facultatif. Donc les obligations qui sont celles qui restent sur les entreprises avec la directive CSRD même dans sa version simplifiée reste déterminée et ambitieuse. La question que vous avez ensuite soulevée de la prévisibilité et de l'instabilité que cela peut créer pour les entreprises, c'est une vraie question. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous avons aussi tôt que possible, avec le DADU, permis de donner de la visibilité aux entreprises pour qu'ils puissent se projeter, pour ne pas que cet effort de simplification vienne créer de l'incertitude supplémentaire puisqu'il s'agit bien de les accompagner. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Luc Brault pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Allons droit au but. Qu'est-ce qui se cache derrière ce débat ? Une passion que la France partage avec l'Union Européenne, la fraisaisie normative. Mes chers collègues, Madame la Ministre, disons-le clairement et simplement, la première des mesures de simplification et d'allègement de la charge administrative des entreprises est très simple, c'est de leur apporter de la stabilité, de la visibilité. Bref, il faut que nous arrêtions de danser le tango à l'échelle européenne, un pas en avant, un pas en arrière. Si nous n'avions pas de complexifié aveuglement, nous n'aurions pas à simplifier par paquet omnibus. Nous avons besoin de l'Union, c'est une évidence, pas de débat. Mais sur le terrain, demandez aux chefs d'entreprise ce qu'ils pensent de la Commission. TPE, PME ou groupe international, tous les patrons français vous le diront. On n'a pas le temps de se mettre en conformité avec une règle, qu'une nouvelle norme nous tombe sur les bras. Et encore, ça c'est pour ceux qui ont les moyens soit d'employer un juriste pour assurer une veille dans leur secteur, soit de gaspiller du temps et de l'énergie à le faire eux-mêmes. Mais tous les autres, il faut le dire, nous avons une forme de précarité administrative et juridique chez beaucoup de nos concitoyens et en premier lieu chez nos chefs d'entreprise. Et ça en devient presque viscéral. Certains ont la boule au ventre chaque jour à cause de ça en se disant « mais à quoi je ne pense pas ou qu'est-ce qui va me tomber dessus demain ». C'est pareil pour tous les patrons des pays de l'Union, me direz-vous. Mais ajoutez-y notre penchant bien français pour le bavardage législatif et la sur-transposition des directives européennes. C'est la cerise sur le gâteau ou plutôt la goutte qui fait des bordels vases. Pourtant, l'Union européenne nous est essentielle, je le redis, pas de débats sur le sujet. Elle nous apporte une stabilité politique dans un monde toujours plus flou et frénétique. Mais la Commission doit asseoir cette stabilité dans son travail normatif en conciliant harmonisation européenne et ambition collective, et non en ajoutant de la frénésie à la frénésie. Donc je crois, Madame la Ministre, que le premier message que nous devons porter auprès de l'Union pour l'avenir, c'est un appel à un changement de logiciel, de culture, et pourquoi pas inspirer de celle du Sénat, de notre assemblée, pour une culture de la sagesse normative. Pour que la priorité des priorités, ce soit simplement d'agir plus raisonnablement, plus connecté au terrain, au lieu de faire de manière précipitée quelque chose qu'on cherche régulièrement à détricoter, ensuite de manière maladroite. Ceci ne doit pas empêcher d'agir avec réactivité, au contraire. Nous gagnerions en souplesse et en perspective sur le temps long pour apporter stabilité et visibilité à nos entreprises et PME. Car je crois sincèrement que c'est la première des préoccupations de nos patrons, savoir ce qui se passe après demain pour choisir comment investir demain. Le résultat est là. Les chiffres ont été dits PIB, innovation, production industrielle. Si nous les Européens ne faisons rien, nous condamnons notre union à une lente agonie. Et c'est certain, ce sont les propos de Mario Draghi en date du 9 septembre dernier lorsqu'il a rendu public son rapport sur la compétitivité européenne. A la suite de ce constat, la Commission nous dévoile en début d'année 2025 une feuille de route afin de réduire le retard économique de l'Union européenne. La simplification des normes, l'allègement des charges administratives pesant sur les entreprises est l'une des priorités de cette feuille de route. La Commission propose donc de revenir sur des normes européennes adoptées ces dernières années afin de simplifier les règles auxquelles sont soumises les entreprises. C'est un meculpa qui ne dit pas son nom, mais faisons-le avant qu'il ne soit trop tard, le plus rapidement possible et principalement pour nos petites et moyennes entreprises. Encore une fois, dans un contexte international marqué par d'importants bouleversements, le retour de la guerre commerciale, il est impératif de manier réactivité et stabilité pour nos PME. Il en va de notre compétitivité, de notre indépendance et de notre souveraineté. je tiens ici à défendre que simplifier nos normes ne signifie pas sacrifier nos objectifs, notamment en matière d'écologie, ça doit rester notre priorité. Je crois même au contraire que si nous agissons au départ de manière moins précipitée, plus proche de la réalité des acteurs économiques et des territoires, nous y gagnerons en termes d'efficacité économique, acceptation sociale et atteinte de nos objectifs qui doivent rester ambitieux. Alors je vais vous poser deux questions Madame la Ministre. Comment la France s'adaptera-t-elle aux mesures de simplification qui seront, je l'espère, adoptées à l'échelle européenne ? Et pouvez-vous nous affirmer qu'ici ensuite, la France sera le garant d'une certaine forme de sagesse normative auprès de la Commission pour apporter visibilité et stabilité à nos entreprises ? Merci cher collègue. Madame la Ministre, Répondrez-vous à ces deux questions ? guide notre action dans cet effort de simplification et c'est pourquoi au ministère de l'économie et des finances sont reçus très régulièrement les entreprises concernées par ces réglementations pour les consulter sur les positions à tenir. Et pour répondre à votre question sur la transposition de ces directives de simplification, nous veillerons bien sûr à ne pas complexifier, à ne pas sur-transposer et à nous assurer que l'effort de simplification est bien ici dans le droit français et qu'il bénéficie à nos entreprises. Votre deuxième question sur la sagesse, j'y répondrai peut-être avec un exemple. Nous ne nous interdisons pas, nous sommes d'ailleurs les seuls sur la directive dont je vais vous parler, à remettre en cause des textes dont nous ne verrions pas l'utilité. C'est le cas pour FIDA. FIDA c'est de nouvelles règles sur les données financières des clients. Nous sommes seuls à avoir cette position mais nous nous battons pour supprimer cette directive parce que nous n'en voyons pas l'intérêt. Nous ne nous voyons pas à l'intérêt suffisant au regard du coût de la lourdeur d'allongement de trois à huit heures des procédures, pour ne prendre qu'un exemple, pour les entreprises. Et donc nous plaidons purement et simplement pour sa suppression. Donc nous savons le faire quand il est nécessaire. Merci Madame la Ministre. C'est bon chers collègues, je continue. La parole est à madame Pascal Gruny et ce pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Européennes, chers collègues. La Commission Européenne a dévoilé récemment son agenda de simplification et un premier programme de travail pour 2025. Je voudrais insister sur le volet agricole de cette démarche. La communication Vision Agriculture 2040 de la Commission comporte quatre grands axes de simplification qui font suite aux quelques mesures actées l'année dernière face à la colère du monde agricole. Certains points méritent que l'on s'y penche. Tout d'abord, la Commission souhaite mettre en place des outils simplifiés d'aide aux revenus. L'empilement actuel des dispositifs ouvrant droit à prestations et les conditions kafkaïennes qui leur sont associées font de la déclaration PAC annuelle un véritable cauchemar pour les agriculteurs. C'est non seulement une surcharge administrative indu, car les agriculteurs sont là pour produire mais pas pour administrer, mais cela multiplie en outre les risques d'erreurs déclaratives et donc en bout de course les risques de sanctions. Dans cette catégorie, la communication contient surtout une phrase qui pour moi est essentielle, je cite « il n'appartient pas à l'union de concevoir en détail les pratiques à respecter dans les exploitations », je dirais enfin. La question des contrôles est absolument centrale pour les agriculteurs. Ils doivent être les moins nombreux possibles et il conviendrait de regrouper en une seule visite tout ce qu'il y a à contrôler. Ces contrôles doivent se concentrer non pas sur le respect de tatillon de telle ou telle norme, mais plutôt sur l'analyse des résultats obtenus. Ils doivent être tournés non pas vers la sanction systématique de l'erreur, mais plutôt vers l'accompagnement technique dans la mise en œuvre de solutions efficaces. La Commission entend également promouvoir les nouvelles technologies comme vecteur de simplification. Ce serait non seulement un facteur de compétitivité pour l'exploitation, avec une meilleure utilisation des ressources et un meilleur pilotage, mais cela permettrait aussi des contrôles plus simples et rapides, certaines données étant déjà suivies et enregistrées. Au surplus, il est avéré que l'utilisation d'images satellitaires permet des contrôles surfaciques beaucoup moins invasifs. Un point général me semble important. La simplification ne doit pas seulement viser une administration plus simple des dispositifs. Elle doit avant tout viser une mise en œuvre plus simple sur le terrain pour faciliter à la fois la vie des agriculteurs et l'atteinte des objectifs politiques de la PAC. Attention à ne pas trahir les attentes. L'effet réel devra être très concrètement perceptible pour les exploitants. sinon ce sera un nouveau coup d'épée dans l'eau. Le Sénat restera par ailleurs vigilant à ce que l'on utilise pas les habits de la simplification pour déguiser ce qui sera en fait une nouvelle étape de renationalisation de la PAC, ce que j'avais déjà dénoncé dès juillet 2017 dans mon rapport sur l'avenir de la PAC. Enfin, si cette initiative sur la simplification va incontestablement dans le bon sens, en espérant qu'elle aille vraiment au bout de la logique, se pose aussi la question d'une éventuelle dérèglementation sur certains points. En effet, des règles plus simples à appliquer, c'est évidemment très bien. Mais la réflexion ne doit pas s'arrêter là. En effet, il est nécessaire qu'elle porte également sur le stock de normes qui s'est accumulé au fil des ans et qui n'a jamais fait l'objet d'un véritable bilan coût-avantage. Or, n'oublions pas que le gouvernement américain fait de la dérégulation l'un des axes centraux de sa politique économique. Il est dès lors à craindre que ce mouvement venu d'Amérique exerce une pression concurrentielle sur le reste du monde, qui in fine pèsera sur l'Europe et aggravera encore davantage le différentiel compétitif dont elle souffre. En agriculture, comme dans d'autres secteurs, nous serons alors placés face à un choix que nous ne pourrons plus continuer d'esquiver, déréguler nous aussi ou, si nous ne voulons pas nous y résoudre, nous protéger, que ce soit à l'américaine avec des barrières tarifaires ou à l'européenne avec des barrières non tarifaires qui donneraient enfin véritablement corps aux principes de réciprocité des normes, les fameuses clauses miroirs dont on parle beaucoup mais dont on voit peu la couleur. Au vu du contexte actuel, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous faire état des réflexions nationales et européennes que vous menez sur le sujet ? Pour conclure, mes chers collègues, le monde agricole a montré au fil des années son incroyable résilience. Toutefois, la pression exercée par les tensions géopolitiques et les crises récentes, les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes et les conséquences des tendances structurelles emmenosent la viabilité. Dès lors, donnons à nos agriculteurs les moyens de faire leur métier sans entraves. C'est à ce prix qu'ils pourront réellement assurer notre autonomie alimentaire et notre indépendance stratégique. Il est urgent d'agir. Merci pour votre attention. Madame la Sénatrice, pour ce qui est de l'agriculture, la philosophie sera la même. Pour les détails, je préfère m'en remettre à la ministre de l'Agriculture. Mais de trouver ce juste équilibre entre le quotidien de nos agriculteurs, je sais que Madame la Ministrie est très attachée. Elle a beaucoup porté un projet de loi qui avait été pris un peu de cours par par l'époque précédente. Pour que nous puissions apporter des réponses très claires à nos agriculteurs, nous puissions les accompagner. Et donc la même philosophie sera la nôtre, celle de simplifier en préservant les objectifs qui sont les nôtres d'un point de vue du pacte vert notamment, mais bien accompagner les agriculteurs qui sont ceux qui nourrissent notre pays et qui font un métier très noble et très important pour notre nation. Merci Madame la Ministre. Allez-y. Madame la Ministre, moi je vais me permettre juste d'ajouter une chose, c'est que moi j'ai toujours peur quand on dit qu'on va simplifier. Donc je dirais à les agriculteurs, ils veulent pas qu'on leur rajoute. Donc c'est surtout ça mon message, simplifier, voilà, sans en ajouter, et simplifier déjà ce qui a été fait précédemment. Merci. Et la parole est à notre collègue Madame Nadejavé pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et ce pour six minutes à vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Il nous faut, oui, simplifier, mais selon toujours deux impératifs, simplifier sans déréguler, simplifier sans complexifier, Alors que le texte relatif à la vie économique reprend à l'Assemblée nationale ou encore un millier d'amendements, il me paraissait utile de le rappeler en introduction, appliquons déjà les règles existence de façon homogène en prenant le temps de les expliquer, les accompagner, de les évaluer. Formons pour se faire celles et ceux à qui elles se destinent avant de faire le procès de leur non ou de leur mauvaise mise en œuvre. Préservons les relations entre nos administrations et les usagers avec notre appareil productif, avec moins de documents et plus de proximité, moins de défiance et plus de confiance. L'excès de normes, leur imprévisibilité, leur complexité pèsent négativement sur l'activité de nos entreprises, sur notre économie. Soit, mais il existe aussi un autre volet qui n'est pas suffisamment abordé, il s'agit de la souffrance au travail et du sentiment d'inutilité, le découragement des équipes que cela génère. La France se classe au deuxième rang des pays où la bureaucratie est la plus complexe. Dans mes récents travaux sur cette problématique, de nombreux témoignages m'ont été adressés tels des appels au secours. Il faut arrêter de légivérer sans cesse. Tout change en permanence. C'est trop dur pour nous. Ma directrice des affaires financières devient folle. Les normes que nous édictons emportent des conséquences sociales. Tous les secteurs attendent de nous des réponses, en France et en Europe. Une forme de sobriété. Aussi, je le dis au préalable, je recrète le choix du rejet du test PME à l'Assemblée nationale. Tout ce qui permet d'éclairer nos décisions et ses conséquences doit être renforcé sur le plan économique et budgétaire environnemental aussi. Il en va au sens pro de notre responsabilité. Hier, à la Maison du peuple de Brest, je défendais d'ailleurs une systématisation des études d'impact, de même que la mise à l'ordre du jour de la motion de censure constructive proposée par François de Rugy en 2015. Aussi, je défends le rétablissement du test PME, tout comme j'ai soutenu la mise en œuvre du test CRSD, pour que les reportings soient finalement praticables au sein des États membres. Après l'inversion de la courbe du chômage, après l'inversion de la courbe des émissions de CO2, soyons déterminés à inverser la courbe ressentie comme exponentielle de la complexité. C'est ce que vous avez proposé, Messieurs Rietman, Moga et Devinas, dans un travail sénatorial remarqué. Simplifié, ce n'est pas que numérisé, c'est aussi humanisé. Mais je reviens au cœur des débats organisés ce soir à la demande du groupe Les Républicains. Dans un document publié il y a deux semaines, le Conseil de l'Union Européenne a dévoilé ses positions sur la proposition de directive visant à amender la CS3D, le règlement taxonomie et la CSRD présentée par la Commission dans le cadre du paquet Omnibus en début d'année. Les deux positions apparaissent comme très proches. Objectif, permettre aux 27 États membres de trouver un compromis avant l'été. Les eurodéputés ont quant à eux eu un premier échange à ce propos en commission juridique du Parlement européen le 23 avril dernier. De grandes divergences existent cette fois entre les groupes sur le reporting de durabilité, sur le devoir de vigilance, alors que, je l'ai rappelé, le calendrier est plutôt serré. Plusieurs points de vigilance ont notamment pu être exprimés par le groupe Renew. Tout d'abord, attention à ce que la simplification ne soit pas synonyme d'un abandonnement de nos ambitions, notamment climatiques. Il est aussi demandé que ce soit maintenu la double matérialité dans la CSRD. Celle-ci favorise des rapports de durabilité plus approfondis et pertinents, et alors que dans le même temps, dans le contexte mondial bouleversé que nous connaissons, la Chine à Cantel, elle, annonçait qu'elle allait l'utiliser avec un seuil plus bas que 1000 salariés. Sur les questions de l'audit, Pascal Canfin a pu défendre sa nécessaire simplification alors que de nombreuses plaintes ont été formulées vis-à-vis de ses déclinaisons pratiques. Il s'est par ailleurs opposé à la suppression de l'harmonisation du régime de la responsabilité civile dans le cadre du droit de vigilance. Enfin, il a été défendu la préservation d'un équilibre entre les deux côtés de la chaîne de valeur. Alors que 90% des fournisseurs des grandes entreprises ont moins de 1000 salariés, si le périmètre d'application est trop limité, alors les grandes entreprises ne pourront pas obtenir les données dont elles ont besoin pour se conformer. En conclusion, il sera de toute façon nécessaire de porter une attention toute particulière à l'écriture des guides de cadrage. Comme pour la commande publique, le temps d'adaptation et la sécurisation juridique sont primordiaux et c'est ça le gage de notre réussite. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, je vous remercie pour cette intervention. Peut-être réagir sur un point particulier, c'est la question du test PME, parce que nous sommes favorables à ce type de dispositif, le gouvernement l'est. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup consulté, nous consultons d'ailleurs toujours régulièrement, et je sais que la délégation c'est notorial aux entreprises aussi, pour pouvoir S'assurer que tous ces efforts sont faits en faveur de nos entreprises et dans ce débat là, la question du test PME est un outil que nous jugeons utile. Il y a encore quelques étapes sur le PGA simplification, je pense notamment à la CMP qui pourront nous permettre de voir si nous arrivons à le rétablir, mais il nous semble que c'est une bonne disposition comme vous l'avez mentionné. Merci, cher collègue, c'est bon. La parole est maintenant à monsieur Michel Massé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen et ce pour cinq minutes. A vous, cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est une réalité. Nos normes sont trop nombreuses, peu lisibles, coûteuses pour nos entreprises qui en souffrent énormément. Notre jardin normatif à la française s'est transformé en une jungle hostile. Cette dynamique présente un enjeu de taille pour notre économie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe est au tournant d'un réagencement de l'ordre économique mondial. Une révolution copernicienne va être menée à l'échelle européenne pour alléger et simplifier la charge administrative qui pèse son entreprise. Dans ce contexte, la présidente Van der Leyen a placé dès juillet 2024 la simplification au centre de son deuxième mandat, avec l'objectif d'ici 2029 de réduire de 35% la charge administrative pesant sur les PME. À cet effet, l'année 2025, et structurer autour d'un programme de travail centré sur la compétitivité et des mesures à la matière qui ont été lancées en début d'année. La diminution de la charge administrative doit servir à renforcer la productivité qui fait tant défaut à l'Union européenne et à supprimer les normes qui paralysent nos entreprises. Alors, trois éléments. Trois éléments expliquent à mon sens cette paradisie. l'accumulation et les modifications fréquentes de la législation européenne qui engendre des chevauchements et des incohérences. Ensuite, la transposition du droit européen crée des différences qui alimentent une concurrence déloyale au sein du marché unique. Par exemple, en Lotte-Garonne, comme ailleurs, ça a été cité par ma collègue tout à l'heure, la sur-transposition des normes dans le secteur de l'agriculture, du bâtiment, du transport, ou autre pénalise les entreprises locales. Mais de tout cela, certainement, on en reparlera prochainement. Enfin, la réglementation européenne est plus lourde pour les PME et ETI que pour les grandes entreprises. En faisant le choix d'être proactif ou de proaction sur la simplification, Administrative, la Commission européenne prend en effet le parti de mettre le droit européen au service d'une politique de croissance. L'adoption des textes à venir pourrait représenter une économie potentielle de 6,3 milliards d'euros sur l'éco-administratif et une capacité d'investissement supplémentaire de 50 millions d'euros. Sur le plan de la méthodologie, ces initiatives doivent intégrer de meilleurs outils d'évaluation, de pilotage et de contrôle en se plaçant du point de vue des entreprises. Par exemple, en 2019, l'Union européenne a publié plus de 13 000 actes normatifs contre 3 000 aux États-Unis. Cet écart gigantesque montre bel et bien que l'Europe est atteinte d'une bureaucratie aiguë. Alors, pourquoi cet échec ? À mon sens, c'est parce que l'Union européenne ne dispose pas d'un cadre d'analyse des coûts et des bénéfices de nouvelles normes qui permettrait de s'interroger réellement sur leurs portées et leurs effets. Face à ce diagnostic, plusieurs initiatives ont été prises ces derniers mois pour mieux évaluer l'incidence des règles européennes existantes et la compétitivité européenne. Cela fait écho à des dispositifs adoptés par notre assemblée dans le cadre de la proposition de loi Rietman qui visait notamment à rendre obligatoire les tests PME. De tels mécanismes répondent à une logique claire. Simplifier la vie économique au service s'accroissance. Toutefois, ces initiatives devront nécessairement concilier la libération entre potentiels économiques avec la préservation d'un modèle social et environnemental européen. C'est le dernier point sur lequel je souhaiterais m'attarder. À mon sens, la simplification ne doit pas se confondre avec la régulation de l'économie. Pour remporter ce défi, l'UE doit aussi s'appuyer sur les atouts de son modèle social et sur sa réponse originale et forte au défi de la transition écologique. Dans ce souci, mon groupe défend une mondialisation régulier. Sur la base de ces remarques, la France doit veiller à défendre à l'échelle européenne une politique de simplification compatible avec des standards sociaux et environnementaux les plus élevés possible, c'est dans cette démarche que nous éviterons la sur-transposition pour atteindre ces standards ambitieux. Enfin, pour dépasser le cadre de notre débat, ces discussions doivent également questionner nos modes de consommation. En effet, le premier prescripteur de l'économie reste le consommateur, le consommateur qui, par son action, a un rôle de promotion d'entreprises plus vertueuses et d'encourager les circuits courts. Madame la Ministre, qu'en pensez-vous ? Monsieur le Président, Monsieur Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour ces questions. Peut-être pour assurer sur le fait que l'objectif dans le PAC Omnibus que nous discutions, que ce soit la CRD, le devoir de vigilance ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est bien d'alléger la charge sur les plus petites entreprises. Et donc non, l'ambition n'est pas de leur faire porter plus de charge que les autres, bien au contraire. Dans tout cet effort de simplification, c'est vraiment ce qui est en jeu. de maintenir nos objectifs en s'assurant qu'on ne freine pas notre compétitivité, notamment pour les petites entreprises pour qui les obligations sont plus lourdes à porter, c'est évident. Ça me permet de revenir sur cette question de la compétitivité, parce que dans le contexte géopolitique actuel, on entend beaucoup cette question de la dérégulation, vous l'avez mentionné, Et il me semble qu'en Européens, maintenir nos objectifs, ça peut être finalement finalement une opportunité aussi de compétitivité pour nos acteurs économiques. Je m'explique. La question des fonds de pension, par exemple, qui investissent à long terme et qui continuent à prendre en compte les risques environnementaux, fait que l'environnement international qui est le notre aujourd'hui conduit ces fonds de pension de plus en plus nombreuses à confier la gestion de leurs fonds aux gestionnaires d'actifs européens. plutôt qu'américains. Dans l'effort d'équilibre, de recherche d'équilibre qui est le nôtre, il ne faut pas oublier qu'il y a bien sûr des objectifs très positifs et compétitifs avec les objectifs qui sont les nôtres en matière de responsabilité sociale et environnementale. Merci Madame la Ministre.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un débat très intéressant que nous avons ce soir et je tiens à remercier mes collègues du groupe Les Républicains de nous permettre d'échanger sur les initiatives européennes en matière de simplification et d'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises, même si le terme simplification peut des fois poser question. Je tiens tout d'abord à saluer la proposition de législation dite Omnibus. Ce paquet vise notamment à alléger les contraintes pesant sur les entreprises européennes engagées sur la voie de la transition écologique. Son ambition est de simplifier la publication d'informations en matière de durabilité, de devoirs de vigilance et de taxonomie. Elle doit aussi faciliter les activités commerciales des petites entreprises à moyenne capitalisation. Ainsi, il sera possible de réduire les charges administratives et réglementaires tout en maintenant les objectifs de transition écologique. Cette initiative va dans le bon sens et c'est heureux. Notons que cette initiative fait suite à deux rapports, rapports que j'ai déjà évoqués lors d'un débat préalable au Conseil et qui ont souligné la perte de vitesse de l'industrie européenne par rapport à celle de la Chine ou des États-Unis. Il s'agit du rapport d'Enrico Letta d'avril 2024 et celui de Mario Draghi de septembre 2024. La législation Omnibus vient donc permettre une traduction concrète à certaines des recommandations de ces deux rapports. Par ailleurs, le discours simpliste et anti-européen que nous entendons lors de chaque campagne d'élection européenne réside souvent dans le fait que les mots de nos entreprises proviennent de l'Europe. Effectivement, permettez-moi de rappeler que la France n'est pas la dernière à faire de la sur-transposition. Les exemples, notamment en droit du travail, sont nombreux. On peut préciser que la France a souvent ajouté des protections supplémentaires pour les travailleurs, allant bien au-delà des exigences minimales des directives européennes. Cela peut rendre le marché du travail moins flexible et également augmenter les coûts pour les employeurs français. D'un point de vue environnemental, la France est là aussi trop souvent dans la sur-transposition. Il suffit de regarder les contraintes lourdes qui pèsent sur nos entreprises agricoles par rapport à celles des autres États membres, et cela a été rappelé précédemment. Enfin, la réduction des délais administratifs est aussi un levier crucial pour améliorer la compétitivité des entreprises. En France, plusieurs types de délais administratifs peuvent être optimisés pour créer un environnement plus favorable aux entreprises. Le processus de création d'une entreprise peut prendre plusieurs semaines, voire mois. notamment en raison des délais liés à l'enregistrement auprès des différentes administrations comme le crève du tribunal de commerce ou l'URSAF. Il en va de même pour l'obtention de certains permis de construire ou des licences d'exploitation. De plus, les entreprises doivent souvent attendre plusieurs mois pour obtenir des remboursements de TVA, des crédits d'impôt-recherche ou des aides sociales. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, la réduction des délais administratifs est essentielle pour améliorer la compétitivité des entreprises en France. En simplifiant et en numérisant les procédures, en harmonisant les délais à l'échelle nationale et en favorisant une meilleure coordination entre les administrations, il est possible de créer un environnement plus favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Pour conclure, Madame la Ministre, les initiatives prises récemment vont pour notre groupe dans le bon sens. Mais il faut poursuivre dans cette voie, car les perspectives économiques sont malgré tout obscures dans le contexte ciopolitique que nous traversons. Merci pour votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour ces différentes questions et ce point de la sur-transposition que vous avez justement pointé. Peut-être pour vous y répondre avec quelques exemples récents, le premier dans le projet d'addu que je mentionnais tout à l'heure, nous avons non seulement transposé le fait stop the clock, arrêter, gagner du temps sur la mise en place des obligations des différentes directives, fidèle à ce qui a été décidé en européen, mais nous sommes allés plus loin. Nous avons décidé de lever l'obligation pénale des dirigeants que nous avions introduit dans le droit français, qui n'était pas une obligation au niveau européen, qui était au choix de chaque gouvernement et que nous avions décidé d'appliquer en France. Nous avons pris conscience de ce point que vous mentionnez et nous avons pris des décisions fortes en la matière. Sur les textes à venir, pour vous parler d'un texte que je connais bien, qui est le projet de loi Résilience, qui était dans cet hémicycle il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons fait, ou en tout cas j'ai fait une priorité de mon action avec ce texte, de ne pas sur-transposer, pour s'assurer qu'on est sur une harmonisation maximale au niveau européen. Il s'agit de la compétitivité de nos entreprises, bien sûr, de ne pas avoir des règles différentes entre chaque état membre et j'y veille avec fermeté sur ce texte-ci. la parole est maintenant à notre collègue Marion Ganales pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Simplifier oui, mais simplifier ce n'est pas renoncer. Il paraîtrait pour le moins contradictoire de multiplier des discours de souveraineté européenne tout en s'alignant sur d'autres normes que les normes européennes, à savoir des normes américaines ou chinoises. Il n'y a pas de puissance productive qui n'est pas une puissance normative. Je souscris ainsi aux propos d'Olivia Grégoire qui indiquait récemment que ceux qui ne font pas la règle la subissent à terme. Les normes sociales et environnementales apparaissent bien souvent comme des coupables idéales du ralentissement économique. Comment peut-on incriminer des directives qui ne sont pas encore pleinement entrées en vigueur pour justifier d'un ralentissement économique européen alors que le rapport Draghi recommande surtout et avant tout un choc d'investissement à hauteur de 800 milliards d'euros pour combler le déficit de compétitivité dont vous avez déjà parlé madame la ministre. Je m'attarderai principalement sur le devoir de vigilance dans mon propos. au cœur de la récente directive de simplification dite Omnibus, et nous pouvons être fiers d'avoir été, en France, les pionner sur ce sujet. La comptabilité est un miroir de la société, et le miroir, s'il donne une image du réel, est aussi un outil puissant de transformation du réel. Il existe une vraie valeur ajoutée à la norme. Loin de se limiter à sa seule portée technique, elle constitue un puissant outil pour les entreprises au service de leurs marchés passés, ou à venir. J'aimerais couper court à une vision assez binaire qui pourrait émerger de ce débat. Il n'y a pas d'un côté les dangereux bureaucrates accrois à la norme et totalement déconnectés des enjeux et défis des entreprises, et de l'autre les hussards bleu blanc rouge des entreprises qui peuvent apporter une réponse simple à un sujet aussi complexe que l'environnement des entreprises normatifs européens. Simplifier, c'est l'action de rendre plus simple, plus facile. Je ne vous apprends rien par cette définition très sommaire. Cela étant, ceci m'amène à poser une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend compliquer la vie des entreprises ? Dans l'océan actuel d'incertitude économique et géopolitique, les entreprises ont besoin que le cap soit maintenu pour élargir au long terme leur horizon de navigation. Ce qui leur complique la vie, ce sont les allers-retours des décisions qui les impactent. Or, c'est précisément ce stop-and-go qui caractérise la position du gouvernement français sur le devoir de vigilance, dite directive CS3D. Le volte-face de la France est difficilement compréhensible. Ces directives imposent aux entreprises de prévenir et corriger les impacts négatifs de leur activité filiale, partenaire, sur les droits humains et l'environnement. Rien que ça quand 160 millions d'enfants travaillent sur les chaînes de production mondialisées et que la planète partout déborde ou brûle, comme le ditrait justement mon collègue député Dominique Pottier. Il renonçait, saignait les millions de victimes de tous les rannas plazas du monde, alors que nous venons de commémorer les 13 ans de cet effondrement ayant entraîné la mort de 1200 personnes employées employées par les sous-traitants de grandes entreprises du textile. Alors qu'elle devait être transportée en juillet 2026, La récente directive stop the clock est venue acter le report d'un an du devoir de vigilance. Madame la Ministre, le gouvernement français préconisait lui un report sinédier, position pour le moins paradoxale sachant que la France a intégré ce devoir de vigilance dans son droit national dès 2017 et que le 30 novembre 22, le gouvernement qualifiait encore notre pays de pionner en matière. Alors qu'est-ce qui fragilise les entreprises ? La directive en elle-même ou les vols de phase successifs quand les entreprises souhaitent un cap et une stabilité des règles ? La Commission européenne, dans son étude d'impact préalable, affirmait clairement que le devoir de vigilance contribuait à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Il est possible de simplifier la vie des entreprises sans porter atteinte à l'objectif poursuivi et sans délai supplémentaire car c'est le sens de l'histoire. Pour cela, il aurait fallu agir sur l'acceptabilité des nouvelles réglementations par les entreprises elles-mêmes. Ne pas les laisser donc seules face à ces nouvelles préconisations et motiver toute la chaîne d'accompagnement des entreprises pour venir leur expliquer qu'elles passeraient très vite du décryptage à l'avantage compétitif. La mise en œuvre de certaines normes a un coût, mais le coût social, écologique et de l'impréparation pour les entreprises sera plus lourd encore. Madame la Sénatrice, je vous remercie pour ces différentes questions. Peut-être pour vous répondre plus précisément sur ces 3D. Vous le savez, la France a été pionnière en la matière du devoir de vigilance. Et la question qui nous a occupé dans l'effort de simplification et qui nous occupe encore, la position de la France est claire là-dessus, c'est de ne pas revenir en arrière, mais d'avoir un cadre qui permet d'être aligné avec le droit français et notamment au niveau du seuil de salarié. Le droit français met ce seuil à 5000 salariés. Oui, c'est ça. Alors que la directive européenne prévoyait de la baisser à 1000 salariés. Mais pour que justement on soit plus prédictif pour nos entreprises et que nous ayons cette stabilité, nous plaidons pour que la directive puisse être le plus fidèle possible à ce qui a déjà été mis en place ici, en France. Merci. Vous voulez reprendre la parole ? une position courageuse et anticipatrice sur quelque chose d'essentiel qui vise à quand même conforter les droits humains et donc l'exploitation aussi quand même de beaucoup de personnes dans le monde, pourquoi la France, d'un coup, a reculé en demandant ce report synédié du devoir de vigilance ? Je ne m'explique toujours pas Ce retour en arrière, espérons que ce recul permettra de prendre de l'élan et pas du retard sur le devoir de vigilance. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. En septembre dernier, le rapport Draghi lançait un cri d'alerte. Depuis 20 ans, l'économie européenne décroche. Face aux États-Unis et à la Chine, notre productivité, notre capacité d'innovation s'effondre. La tendance ne faiblit pas. Au contraire, si rien n'est fait, selon Mario Draghi lui-même, l'Europe est condamnée en l'antagonie. Je crois qu'il est utile de le répéter à l'envie. Si rien n'est fait, l'Europe produira toujours moins de richesses, disposera de moins en moins de ressources et sera impuissante à relever les défis démographiques, sociaux, militaires, environnementaux, migratoires et technologiques de notre temps. Face aux offensives commerciales américaines, aux surcapacités et aux dumpings chinois, face aux investissements massifs qu'existe notre sécurité et notre transition, il n'y a plus de temps à perdre. Restaurer la compétitivité européenne est un enjeu existentiel. Beaucoup reste à faire, mais il est une cause profonde de l'asphyxie de nos entreprises qui nous appartient de traiter rapidement. Le fardeau réglementaire, fruit de nos propres excès législatifs, est bureaucratique. Chaque année, selon l'Eurostat, il coûte 150 milliards d'euros aux entreprises européennes. Ces dernières années, ce fardeau n'a cessé de croître. De 2019 à 2024, l'Union a produit plus de 13 000 textes, soit plus du double, de ce qu'ont généré les États-Unis. Et l'administration Trump s'apprête à creuser davantage ses décors en annonçant une vague de dérégulation sans précédent. Dans l'énergie, la finance, l'intelligence artificielle, les télécoms, la défense, le spatial ou les biotechnologies, les défis sont immenses. Soyons lucides. Jamais nos entreprises ne pourront les relever si nous ne simplifions pas radicalement nos cadres réglementaires. Après des années de surréglementation méthodique, l'Europe semble enfin prendre la mesure de l'urgence. Depuis 2022, le principe du one-out s'applique. Pour chaque nouveau surcoût imposé par une norme, d'autres normes doivent être supprimées à coéquivalent. Depuis 2023, chaque analyse d'impact doit intégrer un contrôle de compétitivité. Depuis 2024, l'objectif est fixé. Réduire de 25% la charge administrative sur les entreprises et de 35% pour les PME. La Commission admet désormais que certaines législations, notamment celles issues du Green Deal, où les objectifs environnementaux sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, sont allés trop loin. Car si les objectifs étaient louables, ils ont aussi engendré des monstres administratifs déconnectés des réalités économiques. Leur révision, parfois avant même leur entrée en vigueur, en est la preuve. à travers la boussole pour la compétitivité, les paquets Omnibus, vous l'avez précisé, et la révision des tests sur le reporting de durabilité, la taxonomie des investissements ou le mécanisme d'ajustement carbone sont des actes positifs. Nous saluons également l'attention portée dès cette année au statut des entreprises intermédiaires, au cadre d'investissements ainsi que les simplifications promises dans l'agriculture, la défense, la chimie, le numérique et l'industrie des carbonés. De façon plus générale, la volonté de passer en revue l'intégralité de l'acquis communautaire est une initiative salutaire, tout comme la mise en place d'un cycle annuel d'évaluation de la législation au sein de chaque portefeuille de commissaire, associant systématiquement les entreprises. Cependant, cette dynamique doit s'inscrire dans la durée. La simplification ne doit plus être l'exception, mais devenir un réflexe permanent de notre culture législative et réglementaire. Il nous faut même aller plus loin, poser ouvertement la question de la dérèglementation. Non seulement simplifier, mais aussi questionner l'utilité même de certaines normes. Certaines doivent être corrigées, d'autres tout simplement supprimées. Madame la Ministre, avec vos collègues en charge des entreprises, votre responsabilité est déterminante. Les attentes de nos entreprises sont immenses. Elles aspirent à retrouver leur liberté d'innover, de produire, de créer de la valeur et de l'emploi. Dans un monde où la croissance n'est plus notre monopole et où la pertinence réglementaire façonne désormais la puissance économique. Les ministères en charge des entreprises sont au cœur de la tourmente. Mais ils doivent être tournés vers ce redressement. Par vos actions, la France peut adresser un message clair à ces entreprises. Celui de la confiance retrouvée est d'une ambition renouvelée pour notre compétitivité. Si demain vous témoignez de cette ambition, vous pourrez compter sur le soutien sans faille des sénateurs de la Commission économique, des sénateurs de la délégation aux entreprises et plus généralement des sénateurs d'utilité économique. Madame le ministre, ne les décevez pas. Merci de votre attention. Madame la Ministre, essayez de ne pas décevoir M. Pernod. Je n'essaye pas, je le fais. M. le Président, M. le Sénateur, peut-être très rapidement sur le synédier, puisque je n'ai pas pu re-répondre tout à l'heure, mais il s'agissait bien de se laisser le temps d'aboutir sur notre position pour le devoir de vigilance, mais pas de reporter ad vitam et ternam. C'était pour ça qu'il y avait eu ce terme-là dans le papier auquel vous faites les références. Je passe sur la question qui vient d'être posée parce que vous avez remis au centre du débat, et ça a été mentionné aussi un peu plus tôt et j'ai pas eu l'occasion encore de m'exprimer sur cette question, la question de l'investissement. Parce que simplifier c'est bien mais ça ne suffira pas, on est bien d'accord pour gagner en compétitivité. Et donc pour donner confiance à nos entreprises sur notre ambition, notre détermination à les accompagner pour qu'elles soient les fers de lance de notre politique d'innovation notamment, je vais prendre un exemple, un secteur qui me tient à cœur, c'est celui de l'intelligence artificielle. Je crois qu'on a fait avec le sommet pour l'action sur l'IA exactement ce que vous m'invitez à faire, c'est-à-dire qu'on a redonné confiance à travers un discours d'abord, celui de mettre la France au cœur de l'intelligence artificielle, Paris, la France entière a été le théâtre de l'IA pendant un certain nombre de jours. On a rayonné à l'internationale, ça a permis de créer une vraie dynamique. Mais au-delà de de ce grand sommet, des images qui ont pu être celles du sommet, il y a eu des actes très forts sur la question de l'investissement. En France d'abord, avec 109 milliards d'euros d'investissement annoncés par le président de la République pour créer l'infrastructure dont on a besoin pour faire tourner nos modèles d'intelligence artificielle. au niveau européen ensuite avec un plan à 200 milliards d'euros public, privé, investiable qui doit nous permettre de renforcer nos capacités à déployer notre propre technologie parce qu'il est fondamental qu'on ait nos propres technologies notamment en intelligence artificielle. On parle beaucoup de souveraineté, cette souveraineté elle se construira ensuite ensuite dans nos entreprises qui sont à la pointe d'une technologie comme l'intelligence artificielle et qui aujourd'hui peuvent nous permettre de ne pas recréer des dépendances à des technologies extra-européennes que l'on subit sur le numérique dans plein d'autres secteurs.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Président de Commission, chers collègues, il est de ces sujets dont on parle avec constance, souvent avec de bonnes intentions, mais qui peine hélas à se traduire par des changements concrets. La simplification administrative en Europe en est un parfait exemple. Car oui, implanter, développer ou simplement maintenir une activité économique en Europe devient un défi croissant. Et cela ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, les chefs d'entreprise, les industriels, les investisseurs dénoncent une surcharge administrative étouffante qui alourdit les coûts, qui brise l'agilité et finit par miner notre compétitivité. En comparaison, nos concurrents, qu'ils soient américains ou asiatiques, souvent chinois, évoluent dans des cadres bien plus souples, souvent plus visibles et par conséquent souvent bien plus favorables à l'investissement. Prenons un simple chiffre, mais qui résume à lui seul l'ampleur du problème entre 2019 et 2024, c'était la précédente commission certes, mais l'Union européenne a produit près de 13 000 nouvelles normes. 13 000, c'est plus du double de ce qu'a adopté sur la même période un pays comme les Etats-Unis. Comprenez-moi, ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une question de lisibilité, de cohérence et d'équation avec la réalité du terrain. Soyons clairs, les directives Omnibus ont le mérite d'exister, c'est un progrès. Mais ce n'est pas encore à la dimension du problème de la productivité et de la création de richesses qui est un impératif. Cela reste timide. Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis élu du Nord et dans le Nord il y a une menace qui plane sur une entreprise importante, Arcelor-Mittal. Et donc trois observations, d'abord la question de l'emploi, 400 familles dans le Dunkerque, 200 à Florence, c'est grave, c'est lourd, c'est un problème économique et social bien sûr. Et puis il y a aussi le refus d'Arcelor d'investir dans la décarbonation. alors même qu'ils sont subventionnés pour sa hauteur de 800 millions sur un projet d'un milliard 7. Et dans le même temps, cette entreprise annonce des investissements aux USA pour un milliard d'euros. Et puis il y a la question de la souveraineté, troisième observation. On a une volonté de réarmer la France et l'Europe, ça a été dit, mais si on n'a pas Une filière acier et une filière aluminium souveraine et autonome, eh bien j'ai bien peur, parce que c'est la même chose pour l'aluminium j'ai bien peur que ces questions du réarmement de la France et de l'Europe restent des mots. Voilà la réalité du monde, cette brutalité. Avec Alain Chantillon, il y a maintenant 3 ans, nous avons commis un rapport sur la concurrence européenne. C'était à l'époque du problème entre Siemens et Alstom, le projet de fusion. Et c'est la vraie compétence de l'Union européenne. Eh bien, les principes qui nous ont été exposés, c'était la concurrence libre et non faussée, le multilatéralisme, le meilleur prix pour le consommateur et puis la norme. Mais ça, c'est un peu le monde d'hier. Ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui, ce sont des États, des empires, des continents. qui aborde l'industrie sous le seul angle de la souveraineté et de la volonté de puissance. Alors Ennoryen Amonté, un laboriaire au XVIIe siècle, disait que la puissance d'un pays se mesurait à son industrie. Ces pays subventionnent leur industrie et utilisent les droits de douane, quoi qu'il en coûte sur le plan financier. voire la bourse aux USA, et il me semble que la réplique de l'Union européenne reste timide. Alors comprenez-moi bien, mes chers collègues, il ne s'agit pas ici de renoncer à nos ambitions environnementales ou sociales, il s'agit simplement de les rendre compatibles avec la réalité économique, A cet égard, il est grand temps d'engager un véritable aggiornamento administratif et fiscal, de penser efficacité,

M. le Président, M. le Sénateur, peut-être pour vous répondre sur cette question de la productivité, de la compétitivité de nos industries. Vous le savez, mon collègue Marc Ferracchi est très attaché à cette question et a eu l'occasion de s'exprimer sur un certain nombre des sujets que vous avez mentionnés, donc un peu la même question que sur l'agriculture. Comme il s'agit d'un secteur particulier, je le laisserai vous développer plus précisément les différents plans d'action qui sont les nôtres, mais nous sommes très attentifs à la situation des entreprises, notamment celles que vous avez mentionnées.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mes chers collègues, Nous avons eu un riche débat demandé fort pertinemment par le groupe Les Républicains, qui ne peut que réjouir le Président de la délégation sénatoriale aux entreprises que je suis. Il prolonge les réflexions conduites au sein de cette délégation sur un double sujet. L'indispensable simplification des charges administratives pesant sur les entreprises d'une part, l'allègement des normes européennes en matière de responsabilité sociale des entreprises d'autre part, Les deux sujets se conjuguent et s'alimentent naturellement. Une leçon doit être retenue de cette séquence normative. Qui trop embrasse, mal étreint, disaient des jarablais. C'est-à-dire que celui qui veut entreprendre ou faire trop de choses à la fois risque de ne rien réussir. Nombreuses sont les initiatives européennes à être justifiées dans leurs principes. mais elles sont élaborées en silos et s'adressent toujours aux mêmes opérateurs économiques, les entreprises. Celles-ci ploient sous l'empilement des normes, elles y voient à juste titre une menace pour leur compétitivité, une entrave à leur croissance, voire même un risque mortel. Si au lieu de se précipiter dans l'accumulation des normes, la Commission européenne avait procédé pour chacune d'entre elles à un test PME approfondi, nous n'en serions pas là. Heureusement, comme certains l'ont souligné, la Commission européenne n'a eu d'autre choix que d'entendre le désarroi des entreprises. Pour stimuler la compétitivité, la déclaration de Budapest du 8 novembre 2024 du Conseil européen lance une révolution en matière de simplification afin de réduire d'au moins 25% la charge administrative des entreprises, seuil porté à 35% pour les PME. C'est une révolution comparable à celle préconisée dans le rapport que j'ai présenté à la délégation aux entreprises en juin 2023 et reprise en partie dans le projet de loi simplification en cours d'examen au Parlement, avec l'obligation préalable d'un test dans les entreprises pour toutes nouvelles normes les concernant. À l'occasion de ce Green Deal, la Commission européenne a fait des choix qui auraient dû être ceux des États et des entreprises. L'exemple le plus choquant a été la décision d'arrêter la production de moteurs automobiles thermiques fixés à 2035 dans toute l'Union européenne. Ni les États, ni les entreprises n'ont été consultées. L'étude d'impact était pour le moins légère. Les conséquences, en revanche, terriblement lourdes. La Commission européenne doit se cantonner à fixer des objectifs. Elle outre-passe ses prérogatives quand elle se substitue aux États au mépris du principe de subsidiarité et impose un choix technologique aux industriels au mépris de la liberté d'entreprendre. que l'on ne s'y méprenne pas. Oui, la transformation profonde des activités économiques est nécessaire, car la décarbonation de notre production est indispensable. Cependant, reconnaissons que les différentes directives et règlements européens adoptés depuis 2019 dans le cadre du Green Deal imposent aux entreprises européennes une charge de travail administrative significative pour un coût non négligeable. Nous l'avons souligné dans un rapport de la délégation aux entreprises consacré à la CSRD dès février 2024, dont les rapporteurs étaient Marion Canales et Anne-Sophie Romani, relayant les alertes et inquiétudes de nombreux chefs d'entreprise, les ETI particulièrement, mais également les PME impactés indirectement dès lors qu'elles sont incluses dans les chaînes de valeur des grandes entreprises concernées. Non, la méthode, et le rythme n'étaient pas les bons. Le choix européen de publication de données à la fois financières et extra-financières est essentiel pour cerner les enjeux de durabilité les plus significatifs. Il avait toutefois un double inconvénient. Premièrement, il doit s'agir non d'obligations de résultats mais de moyens et proportionnés aux objectifs. Deuxièmement, le coût pour récolter, mettre en forme et publier ces normes est élevé. Les entreprises doivent payer divers prestataires au détriment de leurs efforts consacrés directement au projet de transition. Ce sont ces derniers investissements qui doivent être priorisés afin qu'elles puissent rester compétitives. Les normes environnementales et sociales ne sont pas affaiblies. Et d'ailleurs, elles pourraient ne pas s'appliquer du tout si elles conduisent à la disparition des entreprises concernées. La Commission a désormais une approche plus réaliste du nouveau cadre mondial de la compétition internationale. Ce n'est ni une dérogation ni un démantèlement, mais une approche plus pragmatique, proportionnelle et progressive. C'est l'application de la réalité économique dans le droit. C'est renforcer nos entreprises face à l'offensive américaine et asiatique de dérégulation massive et structurelle, en adaptant nos objectifs de transition climatique au nouveau climat des affaires. Merci. Merci cher collègue. Alors mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu mercredi 30 avril à 15h pour les questions d'actualité. Au gouvernement, la séance est levée. Merci Madame le Ministre.